jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2018

ce matin. Elle se trouve actuellement auprès des agents hospitaliers, des patients et des autorités de Guadeloupe, à la suite du violent incendie qui a touché, comme vous le savez, le CHU de Pointe-à-Pitre, mardi dernier. Nous nous retrouvons donc pour l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. L'examen du texte en première lecture par les deux assemblées a permis, je veux le souligner, de constater des convergences, et même un consensus, sur de nombreux points- preuve en est le nombre d'articles adoptés conformes, 37 au total, dont les articles d'équilibre. La nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a confirmé ce constat, puisque des articles majeurs- sur la vaccination, le tabac ou le tiers payant, par exemple -ont également été votés dans la version adoptée par le Sénat. 2018 engage la transformation du système de santé que le Gouvernement souhaite conduire. Il vient en soutien de la stratégie nationale de santé, dont la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, arrêtera les orientations dans quelques semaines, à l'issue d'une concertation publique lancée début novembre.

Les dispositions relatives à la vaccination obligatoire des jeunes enfants ont fait l'objet, comme je viens de le souligner, d'un large consensus au sein des deux assemblées. Il en est de même de la priorité donnée à la lutte contre le tabac, en portant à dix euros le prix du paquet de cigarettes. À cet égard, le Gouvernement veut réaffirmer sa détermination à agir, à l'échelon national comme à l'échelon européen, pour lutter contre les trafics et la contrebande. La reconfiguration de la taxe sur les boissons sucrées a également été validée comme un outil pertinent de la lutte contre le surpoids, notamment chez les jeunes. Comme le Gouvernement s'y était engagé, les travaux d'expertise avec les industriels du secteur ont été poursuivis, et l'Assemblée nationale a adopté, mercredi dernier, un barème correspondant au souhait, partagé sur toutes les d'une mesure incitative pour les producteurs, mais qui ne pèse pas fortement sur les ménages. Ces trois mesures, auxquelles s'ajoute la prise en charge d'une consultation de prévention des cancers du sein et du col pour les femmes de 25 ans, sont les marqueurs d'une volonté politique forte et transpartisane d'agir en profondeur sur les déterminants de santé. Ce mandat, très clair, donné par le Parlement viendra conforter la construction du plan national et des projets régionaux de santé, élaborés dans le semestre à venir. Nous faisons également le constat d'une très large adhésion du Parlement aux orientations et aux outils proposés pour faire évoluer notre système de santé. L'article 35 du projet de loi donnera possibilité d'expérimenter, de financer et d'évaluer des organisations différentes, dépassant les clivages sectoriels de l'hôpital et de la ville, du soin et de la prévention, et incitant à la pertinence des soins. Enfin, un consensus s'est également exprimé autour de la volonté du Gouvernement de lever les obstacles au développement de la télémédecine. C'est l'un des volets du virage numérique que le système de santé doit prendre et que le Gouvernement impulsera au cours des prochains mois.

Vous avez exprimé au cours des débats votre grande attention à la mise en oeuvre de cette réforme. Je veux redire ici que le Gouvernement entend donner le temps et les moyens nécessaires à cette transformation de grande ampleur. La période de transition qui s'ouvrira le 1 janvier 2018, permettra de faire évoluer progressivement les organisations de travail et de mener un dialogue social de qualité avec les salariés et leurs représentants. Elle n'impose pas de date butoir s'agissant de l'évolution des systèmes d'information. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que l'organisation mise en place permette une évolution graduée et maîtrisée de ces systèmes, dans des conditions de sécurité garanties. Je veux aussi dire son attachement à la reconnaissance, au sein du régime général, de la spécificité de la situation des travailleurs indépendants, de façon à adapter le service qui leur est rendu. Ces points de convergence sont très significatifs. Le Gouvernement, comme l'Assemblée nationale, les a constatés pour se féliciter du travail parlementaire de grande qualité qui a été conduit. Cependant, ils ne peuvent dissimuler des désaccords sur des dispositions essentielles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, raison pour laquelle votre commission des affaires sociales a adopté, hier, une motion tendant à opposer la question préalable et à ne pas débattre du nouveau texte. Le principal désaccord porte- bien évidemment, allais-je dire -sur la baisse des cotisations salariales, en contrepartie d'une hausse de la CSG. L'Assemblée nationale a confirmé son vote de première lecture, en améliorant le dispositif sur des points que vous aviez relevés, notamment sur les aidants ou les artistes auteurs. Cette disposition du projet de loi a été longuement débattue. Je veux rappeler que cette mesure conforte l'assiette du financement de notre protection sociale en étant certainement plus en phase avec l'évolution de notre modèle social. Il s'agit d'une disposition sans incidence sur les plus petites retraites. Et c'est aussi une mesure qui doit permettre d'accroître, de façon substantielle, le pouvoir d'achat de près de 20 millions de salariés et d'alléger les charges des trois quarts des travailleurs indépendants. Un deuxième point de désaccord a trait aux dispositions relatives à la prestation d'accueil du jeune enfant, la PAJE. Vous en avez également beaucoup débattu en première lecture avant de voter la suppression de l'article 26, que l'Assemblée nationale a rétabli en nouvelle lecture. Dans la construction de ce premier PLFSS de la mandature, des choix ont été faits en faveur des familles les plus pauvres, et notamment des familles monoparentales. Ces choix conduisent globalement à augmenter de plus de 70 millions d'euros la dépense en faveur des familles en 2018. Il s'agit d'une orientation forte de l'action gouvernementale, celle de considérer que la politique familiale a une place essentielle dans la stratégie de lutte contre la pauvreté. Pour autant, ces choix ne résument évidemment pas

à l'issue de l'examen par l'Assemblée nationale du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en nouvelle lecture, 38 articles restent en discussion.

comptes sociaux. Outre la trajectoire financière, le Sénat a marqué son accord avec les orientations proposées en matière de santé : le développement d'une politique de prévention, notamment en matière vaccinale, une démarche d'expérimentation en matière de prise en charge des parcours de soins et la promotion de la pertinence des actes et de l'innovation. Sur le RSI, nous sommes attentifs aux conditions de la réussite de la réforme. Nous avons alerté le Gouvernement sur les points décisifs. Je suis convaincu que les travaux des deux assemblées y ont contribué, dans la complémentarité.

mais sur l'augmentation de 1,7 point de la CSG sur les pensions de retraite et d'invalidité. Ce point de désaccord, qui représente 4,5 milliards d'euros, a suffi, à lui seul, pour constater l'échec de la commission mixte paritaire. Nous pensons que les effets collatéraux de l'augmentation de la CSG ne sont pas tous identifiés. Nous exprimons de doutes sur le sens qu'il y a à financer l'assurance chômage par l'impôt. À l'article 26, le Sénat a marqué son désaccord avec les choix du Gouvernement sur la prestation d'accueil du jeune enfant. Alors qu'une réflexion va s'ouvrir sur les objectifs de la politique familiale, cette mesure n'était, à tout le moins, ni impérative ni urgente. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est revenue, pour l'essentiel, à son texte de première lecture, en particulier sur ces deux principaux points de désaccord. Si elle a retenu certains apports ponctuels du Sénat, elle a supprimé d'autres articles, adoptés avec l'avis favorable de la commission en troisième partie. Je pense notamment à l'extension des exonérations de cotisations aux EPCI pour l'aide à domicile, au cumul emploi-retraite des médecins retraités en zones sous-denses ou encore à la durée des contrôles URSSAF. Sur la troisième partie, je voudrais encore signaler deux points : l'Assemblée nationale a revu le barème de la taxe sur les boissons sucrées pour en limiter le rendement supplémentaire, tout en en préservant néanmoins une partie. Sur l'initiative du Gouvernement, les députés ont modifié les tableaux d'équilibre de fin de troisième partie pour tenir compte des votes intervenus au cours de l'examen parlementaire.

Il serait souhaitable que le Gouvernement apporte des précisions quant au détail de l'impact sur les recettes des différents votes intervenus au Parlement. Les règles d'arrondi et la présentation de ces tableaux « à la centaine de millions d'euros près », nuisent à la qualité de l'information apportée. Ces tableaux, qui seront les tableaux définitifs du texte, mériteraient un niveau de détail beaucoup plus important. Concernant l'assurance maladie, l'Assemblée nationale est revenue sur la plupart des évolutions du texte adoptées au Sénat, à quelques exceptions près, par exemple, le développement des modes d'exercice « coordonné », et non seulement « regroupé l'extension de l'accès au dossier pharmaceutique pour les pharmaciens biologistes ou la reconnaissance du rôle des pharmaciens d'officine dans le déploiement de la télémédecine. En revanche, ont notamment été supprimés la mention spécifique de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale chronique dans le champ des expérimentations, la création d'une procédure d'utilisation testimoniale éclairée et surveillée, les ajustements apportés à la régulation du secteur du dispositif médical ... Nos désaccords avec l'Assemblée nationale ne sont pas nombreux, mais ils sont suffisants.

Ainsi que nous le faisons chaque année, et comme nous y encourage le ministre de l'action et des comptes publics, nous allons désormais entrer dans une phase d'évaluation et de contrôle de l'exécution des lois de financement passées. C'est donc une nouvelle séquence qui s'ouvre et qui pourra déboucher, je l'espère, sur une préparation

dont les tableaux d'équilibre des différentes branches et la trajectoire pluriannuelle des comptes sociaux. Le Sénat a marqué son accord, souvent avec enthousiasme, en faveur du développement d'une politique d'innovation-

Malheureusement, un ensemble d'amendements, en particulier l'amendement relatif à la suppression du mécanisme de la CSG sur les pensions de retraite, ont généré un déficit de 7 milliards

de la sécurité sociale et la CMP ne pouvait que constater l'ampleur des différends, en particulier sur la CSG. Et pourtant, nous avons pourtant prouvé à plusieurs reprises que nous étions capables de nous entendre, capables de nous accorder sur la nécessité de protéger les plus faibles. dans le même temps, d'assurer l'équilibre financier du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tout nouveau déficit générera de la dette supplémentaire et nous empêchera de respecter nos engagements européens, rendant, une fois de plus, la parole de la France totalement inaudible. cette dette devra être remboursée par les générations futures, ce qui rend leur avenir incertain. Être en politique, c'est s'engager à construire l'avenir de nos enfants et des générations futures. Produire du déficit est l'exact inverse C'est pour cette raison, mes chers collègues, que la proposition du Sénat sur la CSG n'est pas tenable. Elle l'est d'autant moins que le Gouvernement, à travers l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, a tenu à protéger les plus fragiles en adoptant des mesures en faveur du minimum vieillesse, de l'allocation aux adultes handicapés ou encore en aidant les familles monoparentales. Resituons l'application du mécanisme de la CSG sur les pensions de retraite dans son contexte global. La proposition initiale du Gouvernement sur les exonérations de la CSG cumulées à la suppression de la taxe d'habitation permet à tous les retraités percevant moins de 2 500 euros d'échapper à une baisse de pouvoir d'achat. Je le redis : les personnes âgées dont les revenus sont inférieurs à 2 500 euros ne seront pas impactées, à terme, par la hausse de la CSG. L'effort doit être collectif, mais réparti. Il n'est pas anormal de demander à chacun de participer à hauteur ses moyens. Il reste assurément des ajustements à apporter, et nous en sommes capables,

égard aux débats qui nous ont animés en première lecture, je suis intimement persuadé que nous pouvons y parvenir. Profitons-en pour mettre en évidence l'intérêt du système bicaméral et l'importance du Sénat dans ces débats. À ses détracteurs, je rappelle que ce système est essentiel à un fonctionnement équilibré de nos institutions, à la représentation de nos territoires et à une élaboration apaisée de la loi.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, quelles remarques nouvelles formuler au moment d'aborder cette nouvelle lecture du PLFSS pour 2018 ? Le texte que nous retrouvons ici ne tient que peu compte du travail des sénatrices et des sénateurs.

Pourtant, quasiment chaque semaine, des personnels nous alertent et mènent des actions contre la détérioration de leurs conditions de travail et, de fait, contre la dégradation de la qualité d'accueil des patients. Et, comme si cela ne suffisait pas, la Cour des comptes recommande, dans son rapport sur l'avenir de publié mercredi dernier, de supprimer davantage de lits d'hospitalisation. Une fois de plus, l'argument de la qualité et de la sécurité des soins est invoqué pour restructurer l'hôpital et réduire le nombre de lits, alors que les hôpitaux de proximité ont déjà été supprimés au profit de territoires, ou GHT. Il est certes nécessaire de faire évoluer l'hôpital et ses pratiques. Mais de quelles évolutions avons-nous besoin pour renforcer notre système de santé ? Comment ne pas voir que les demandes demandes croissantes exigées des équipes pour tout codifier nuisent le plus souvent au temps passé près des patients et accroissent le stress des personnels soignants ? Malheureusement, la Cour des comptes, dont on connaît l'influence auprès des gouvernements, aborde la question dans la continuité des propos de la ministre des solidarités et de la santé, selon laquelle 25 % des actes seraient inutiles à l'hôpital. Ainsi, les sages préconisent, par exemple, de diminuer d'un jour et demi l'hospitalisation pour les prothèses de genou ou de hanche. Les patients passeraient ainsi de 5 à 3 jours et demi d'hospitalisation, et tant pis pour les risques de complication et de retour à l'hôpital en urgence ! Or développer l'ambulatoire nécessite d'en créer les conditions en faisant en sorte que les patients soient pris en charge à domicile. Cela passe notamment par des personnels médicaux et paramédicaux en nombre suffisant, ce qui est loin d'être le cas. Dans ce contexte de flux tendu, que veut dire « moins de lits d'hospitalisation » ? Quelles conséquences sur les urgences ? Je vous invite, mes chers collègues, à prendre connaissance

que la présence d'autres professionnels soignants, ainsi que d'un centre de santé public par bassin de vie, permettant un travail pluridisciplinaire. L'implantation de services publics de proximité est également une condition indispensable à l'installation de professionnels de santé. De plus, il est tout à fait dommageable que l'investissement public ne soit pas non plus au rendez-vous dans les facultés de médecine, afin de permettre de supprimer le tout en donnant aux universitaires les moyens d'assurer les tutorats. Comme je l'ai souligné, la majorité La République en Marche a rétabli, pour l'essentiel, le texte du Gouvernement. Ainsi la hausse de 1,7 point de CSG est-elle toujours au menu pour les salariés et les fonctionnaires, mais également pour les retraités et les bénéficiaires de pension d'invalidité, contrairement aux modifications adoptées par le Sénat. La seule nuance concerne le dédommagement perçu par les aidants familiaux au titre de la prestation de compensation du handicap, la PCH, qui ne serait plus considérée comme un revenu du patrimoine, mais comme un revenu d'activité permettant ainsi de bénéficier d'un taux de CSG de 9,2 %, contre contre 9,9 % dans la première mouture du texte. Quelle générosité ! De la même manière, les députés ont adopté un amendement pour compenser la hausse de la CSG pour les artistes auteurs. La future réforme de l'assurance chômage les concernant y est sans doute pour quelque chose. solidarités et de la santé a annoncé le dégel de 150 millions d'euros de crédits pour les hôpitaux. Comment s'en plaindre ?, même s'il faut redire que vous prévoyez une baisse de 1,2 milliard d'euros et que le montant de ces crédits est légèrement inférieur- de moitié ! -à ce que les établissements hospitaliers réclamaient. La seule épidémie de grippe programmée au mois de décembre risque de réduire la portée de ce reliquat. Pour notre part, nous aurions souhaité qu'une partie de cette somme aille à l'hôpital de Bastia, que plus d'un millier de personnes ont manifesté samedi dernier pour sauver. Comment ne pas évoquer la situation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, l'AP-HP, qui a annoncé la suppression de 180 postes non médicaux, en majorité dans les services de santé pour 2018 ? Les comptes du plus grand hôpital français connaîtraient une telle dégradation qu'une baisse du nombre de salariés en CDD principalement dans les services de soins- 101 équivalents temps plein, ou ETP -et parmi le personnel administratif- 49 ETP. Ces réductions drastiques expliquent sans doute les menaces qui pèsent sur deux services de l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil, à l'origine d'une demande de rendez-vous des six sénatrices et sénateurs du Val-de-Marne, toutes sensibilités politiques confondues. En outre, je vous invite, mes chers collègues, à regarder le nouveau documentaire de Raymond Depardon, intitulé, sorti cette semaine, qui montre les symptômes d'un inquiétant virage sécuritaire dans le monde de la psychiatrie. Filmé au centre hospitalier Le Vinatier, à Bron, il met en exergue les conséquences des réductions de moyens, qui entraînent le développement de protocoles standard à respecter, et les réductions de personnels, qui favorisent le recours à la contention. Je le redis avec force, une politique alternative de santé est possible, dès lors que les choix budgétaires sont mis en oeuvre en conséquence. Je ne vous ferai pas l'injure de répéter toutes les propositions de financement que nous avons formulées en première lecture et qui donnent crédit à nos propositions, car je suis certaine que vous les avez encore en mémoire. Cette politique alternative de santé consiste à aller vers un remboursement des soins à 100 % par l'assurance maladie, plutôt que vers un « zéro reste à charge » reposant sur les complémentaires, au détriment des ménages, à avoir un service

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, une nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ? Un exercice dont nous savons qu'il sera écourté et dont l'utilité n'apparaît pas certaine ... Qu'exprimer à ce moment ?

Des regrets, aussi, de voir une discussion interrompue, un fonctionnement de la démocratie qui ne va pas au bout de ses possibilités, sans remise en cause de l'exigence du bicamérisme, mais qui pose toutefois la question des nouvelles lectures pour les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale. Combien de nouvelles lectures ont-elles été conduites jusqu'à leur terme au cours des dix derniers exercices ? Des regrets, encore, à constater que l'Assemblée nationale est revenue, pour l'essentiel, à son texte de première lecture. Ce n'est pas une surprise s'agissant des points forts de divergence, relatifs à la hausse de la CSG ou à l'évolution de la prestation d'accueil du jeune enfant.

la mention spécifique de la prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale chronique dans le champ des expérimentations- au moins, sur ce dernier point, le débat a-t-il été lancé. Quelques satisfactions,

obligation vaccinale, consultation gratuite de prévention du cancer. Ils ont aussi soutenu avec vigilance, en apportant leur part au débat, les mesures d'expérimentations organisationnelles et le développement de la télémédecine. Le texte

à l'utilisation telle qu'elle est définie du produit de la CASA, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, ou à l'alignement des déterminants de l'allocation de base sur ceux du complément familial qui entraîne une baisse de la prestation d'accueil du jeune enfant. Opposition, aussi, au dispositif d'ajustement à la baisse des prix et tarifs des dispositifs médicaux ou à l'évolution du tiers payant généralisé en tiers payant généralisable, pour ne citer que les principaux points.

Le rapport, plutôt explosif, si j'en crois les premières réactions, est celui de la Cour des comptes- il a été évoqué précédemment. Je cite rapidement les grandes lignes du jugement porté sur notre système de santé : des résultats globalement satisfaisants, mais des faiblesses persistantes, des politiques de maîtrise de la dépense trop souvent mises en défaut, des modes de régulation en échec. Une perspective est tracée : donner la priorité aux objectifs de santé publique et de qualité des soins.

au début du mois de novembre, notre chambre a étudié le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, avec l'objectif de tenir le cap, fixé par le Premier ministre, d'un équilibre des finances sociales à l'horizon 2020,

Le Sénat a voté la suppression de la hausse de 1,7 point de la CSG sur les pensions de retraite. Cette mesure n'est pas tenable sur le plan financier et nécessitera qu'une part de la TVA soit réaffectée au budget de la sécurité sociale, afin de compenser le manque à gagner de 4,5 milliards d'euros. s'agit donc d'une perte sèche pour l'État, aggravant notre situation financière nationale. Cette décision nous a mis dans l'impasse ; c'est la raison pour laquelle mon groupe s'était abstenu au moment du vote de ce texte. Lors des débats sur l'article 7 du PLFSS pour 2018, nous avions proposé une solution intermédiaire : maintenir une hausse de la CSG sur les pensions de retraite, tout en la limitant à 1,2 point. L'Assemblée nationale aurait peut-être pu la retenir.

mise en place d'innovations expérimentales, résorption des déserts médicaux et soutien à l'implantation des médecins en zone rurale, simplification des dispositifs devenus trop complexes, anticipation des transformations numériques de la santé, etc. Il est essentiel que nous étudiions ce texte ensemble, représentants de la droite et de la gauche, majorité et opposition, pour assurer un équilibre des comptes de la sécurité sociale d'ici à 2020. de la réforme du financement de la sécurité sociale, le Gouvernement envisage un effort salutaire de limitation de l'augmentation des dépenses de sécurité sociale à 2,1 % sur la prochaine année. C'est un effort d'économie courageux. Il s'agit d'une première étape sur la route d'un équilibre des comptes à l'horizon 2020, malgré les problèmes annoncés de la branche vieillesse.

De manière générale, l'Assemblée nationale a détricoté une bonne partie des mesures que nous avions votées à l'article 7 : fixation du taux de cotisation de solidarité des petits exploitants agricoles, réduction du taux de cotisation vieillesse des artistes-auteurs, etc. Mon groupe regrette que les amendements adoptés en séance par l'Assemblée nationale aient, dans leur quasi-totalité, simplement rétabli la rédaction adoptée en première lecture par cette même assemblée. Si nos collègues députés nous écoutent, telle n'est pas notre vision du débat parlementaire : la loi s'écrit par le concours conjoint de l'Assemblée nationale ... et du Sénat

les mesures de rationalisation et de simplification de la sécurité sociale, le groupe Les Indépendants-République et Territoires partage entièrement la volonté du Gouvernement de simplifier le régime de sécurité sociale français et d'y apporter une plus grande lisibilité.

de penser qu'il est possible d'aller encore plus loin sur ce sujet. Nous avions ainsi déposé des amendements relatifs à la prévention qui n'ont finalement pas été retenus. Nous regrettons par ailleurs que les députés aient supprimé l'article 9 , introduit par notre chambre, qui encourageait le cumul emploi-retraite pour les médecins retraités exerçant en zone sous-dense. Notre orateur de groupe, le sénateur Chasseing, avait d'ailleurs fait remarquer que les deux chambres avaient voté une telle disposition, lors de l'examen de la loi Montagne, pour les zones montagneuses. Il semble donc que cette mesure fasse consensus entre nos deux chambres et soit un outil approprié pour accompagner le renforcement du tissu médical dans les zones sous-dotées. S'agissant enfin des mesures d'adaptation de la sécurité sociale et de notre modèle de santé au monde de demain, mon groupe a été très sensible aux propositions d'expérimentations en faveur de l'innovation dans notre système de santé. Téléconsultation, téléexpertise, téléradiologie : la médecine de demain s'invente aujourd'hui. Il y a quelque temps, à l'occasion d'une semaine de contrôle, nous avions posé la question de la rencontre de la loi et du numérique, en nous interrogeant sur l'encadrement juridique des nouvelles technologies. Cette question s'applique également à la nouvelle relation de la santé et du numérique. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon groupe souhaite que la Haute Assemblée poursuive l'examen de ce projet de loi, selon une démarche constructive et sereine.

nous en arrivons à la nouvelle lecture de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, après un échec de la commission mixte paritaire et une deuxième délibération, avant-hier, à l'Assemblée nationale. M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales propose d'arrêter là la discussion sur les articles restant en navette.

le nombre d'articles restant en navette : 38 seulement. Certes, j'ai bien entendu les arguments avancés par le rapporteur général du Sénat s'agissant des divergences entre les deux assemblées, principalement au sujet de l'article 7. Toutefois, des solutions ont pu être trouvées concernant les bénéficiaires de la PCH, les artistes-auteurs, ou encore les agriculteurs. Dans sa grande majorité, mon groupe pense donc que les

Peut-être pourrions-nous également, à l'avenir, et comme cela a déjà été évoqué et souligné par certains, engager les discussions avec les députés avant même la première lecture, afin d'obtenir un consensus sur les sujets majeurs. Parmi les points d'accord avec les députés, je saluerai tout de même les avancées en matière de politique de prévention et d'innovation- je citerai le passage à onze vaccins obligatoires pour les jeunes enfants, ainsi que les articles 35 et 36 sur l'expérimentation et la télémédecine, autant de points qui vont dans le bon sens.

ce qui concerne le tiers payant généralisé, je partage, à titre personnel- telle n'est pas la position majoritaire de mon groupe -, la position de la ministre des solidarités et de la santé : la réforme, en l'état, n'était pas applicable ; un report me semble être la meilleure solution. Quant aux déserts médicaux, je regrette vraiment que l'Assemblée nationale n'ait pas conservé la proposition du Sénat consistant à exonérer partiellement de cotisations vieillesse les médecins retraités exerçant en zone sous-dense. Il s'agissait, selon moi, d'une solution facilitatrice, incitation à la poursuite de l'exercice médical. Au vu de la désertification médicale frappant tous nos territoires, nous déplorons la décision de rejeter cette proposition. des dispositifs médicaux à domicile, nous regrettons également la réintroduction par l'Assemblée nationale d'un alinéa de l'article 41, supprimé par le Sénat en première lecture, qui prévoit de plafonner le nombre de prestations

Je reste enfin perplexe quant à l'intérêt d'une fiscalité spécifique sur les boissons sucrées et édulcorées. Comme l'a rappelé mon collègue Guillaume Arnell lors de son explication de vote en première lecture, cette comportementale risque de frapper en premier lieu les populations défavorisées. Nous préférerions et espérons encore une ambitieuse politique d'éducation à la santé.

Je rappelle, pour finir, la proposition qui a été faite par le groupe du RDSE en première lecture concernant la généralisation de la vaccination contre le papillomavirus- la ministre a évoqué la possibilité d'un débat sur ce point. Mon groupe y est très favorable et sera attentif aux propositions du Gouvernement dans ce domaine.

Bien sûr, il est tout à fait légitime que nous restions sur nos positions- elles ont été largement exprimées. Des conceptions différentes s'opposent, concernant notamment

méritera une attention toute particulière. On peut se poser des questions quant à la gestion paritaire de l'assurance chômage, compte tenu des

mes chers collègues, nous avons adopté, en première lecture, le premier projet de loi de financement de la sécurité sociale du quinquennat, après plusieurs jours de discussions très riches,

provenant de toutes les travées et de la commission. Nos échanges ont été riches, nourris, précis, sur des sujets parfois très techniques- mon collègue René-Paul Savary vient d'en évoquer un ; ils se sont déroulés dans un climat serein et dans un esprit constructif.

Ces remerciements s'adressent également à nos rapporteurs, qui ont su guider, par leurs précisions techniques, nos réflexions sur l'ensemble des thématiques abordées dans le cadre de ce texte. Évidemment, personne ne s'attendait à ce que la commission mixte paritaire aboutisse- nous l'aurions bien voulu ! -, en dépit du climat que je viens de décrire. La modification de l'article 7 et la suppression de l'article 26 ont empêché le consensus de se former, ce qui peut se comprendre : deux visions différentes se sont affrontées. Le Gouvernement, soutenu en grande partie par sa majorité à l'Assemblée nationale, a souhaité financer un surcroît de pouvoir d'achat à destination des actifs par une hausse de la CSG. C'est l'objet de l'article 7 ce PLFSS. Nous comprenons cette logique, même s'il nous semble qu'un effort supplémentaire de pédagogie aurait été salutaire, notamment auprès des retraités.

de la baisse de la taxe d'habitation- nous avons eu l'occasion de l'expliquer. Il aurait sans doute été possible de trouver une solution intermédiaire, par exemple en lissant cette augmentation sur deux ou trois ans. vous faites un choix et vous l'assumez ; personne ne peut reprocher au Président de la République d'appliquer son programme. Nous espérons désormais que le pouvoir d'achat des retraités sera préservé.

Sur ces deux marqueurs forts de ce PLFSS, l'échec des discussions était donc assez prévisible. Ce qui se comprend moins, en revanche,

Certaines mesures auraient permis d'améliorer l'organisation et l'accès aux soins. Comme l'un de mes collègues l'a rappelé, l'extension de l'exonération de charges sociales aux EPCI organisant un service d'aide et d'accompagnement à domicile

particulièrement touchés par la désertification médicale. Mon intervention ne se veut pas pour autant un réquisitoire à l'encontre de ce premier PLFSS. La navette parlementaire a malgré tout permis de conserver des mesures issues des travaux du Sénat,

La prise en charge de ces publics vulnérables par différents dispositifs peut être simplifiée et gagner en lisibilité ; les bénéficiaires et les services qui les accompagnent ne s'y retrouvent pas tous.

de faire un premier bilan des actions que vous avez engagées. Nous aurons alors plus de temps pour instaurer un dialogue plus en amont, comme cela a été évoqué en commission mixte paritaire.

la motion. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, au terme de la discussion de ce projet de loi, le bilan qu'en tire la commission des affaires sociales peut se résumer à trois séries d'observations, qui recoupent en réalité trois grands groupes de dispositions, sur lesquelles nous nous trouvons, par rapport au Gouvernement et à l'Assemblée nationale, dans des positions bien différentes. Tout d'abord, cela a été dit, une grande majorité des articles du texte ne suscitent aucun désaccord de fond

la taxation des boissons sucrées, la vaccination, les consultations de prévention pour les jeunes femmes, la suppression de l'obligation générale du tiers payant, ou encore les expérimentations visant à promouvoir un véritable parcours de soins et une meilleure efficience des prises en charge. Je ferai une mention particulière sur l'affiliation des travailleurs indépendants au régime général et sur la suppression du RSI. J'avais fait part, en première lecture, de mes réserves sur l'inclusion d'une telle réforme dans un projet de loi de ses interrogations sur la capacité d'une telle réforme à réellement régler les difficultés identifiées ces dernières années, la commission des affaires sociales a choisi de compléter le texte et tenté de l'améliorer. Je constate que, pour une très large part, l'Assemblée nationale a conservé les amendements que le Sénat avait adoptés. Face à ces points d'accord, les points de désaccord, cela a été dit également, se limitent finalement à deux dispositions principales. Si le Sénat a supprimé l'augmentation de 1,7 point du taux de CSG applicable aux pensions de retraite et d'invalidité, c'est d'abord parce que cette nous a paru injuste dès lors que, pour toutes les autres catégories, le Gouvernement a prévu des mesures de compensation. Cette hausse de CSG représente, monsieur Lévrier, 4,5 milliards d'euros de prélèvements supplémentaires sur les retraités. L'exonération de taxe d'habitation, qui ne représente que 3 milliards d'euros pour l'ensemble de la population, ne peut valablement apparaître comme une véritable compensation. Mais au-delà de ce point peu justifiable à nos yeux, cette hausse de CSG nous paraît introduire des éléments de brouillage dans le financement de la protection sociale.

Elle transfère vers l'impôt le financement de risques à caractère assurantiel. Elle augmente la part des prélèvements sur les revenus d'activité dans le financement la sécurité sociale et diminue celle des prélèvements sur la consommation. Il y a donc là un point sur lequel nos deux assemblées ne pouvaient s'accorder. L'autre divergence porte sur les règles d'attribution de la prestation d'accueil du jeune enfant, Cette mesure, peu justifiée au regard de la situation financière de la branche famille, restreint un peu plus le périmètre des bénéficiaires de la politique familiale et a été largement rejetée par notre assemblée. Enfin, une dernière série de dispositions témoigne de désaccords, qui, à mon sens, auraient pu être surmontés, car ils ne résultent en rien de divergences philosophiques ou de fond. Sans doute les délais d'examen extrêmement contraints du projet de loi de le dialogue avec le Gouvernement et l'Assemblée nationale. Je regrette toutefois que certains amendements adoptés par le Sénat, parfois depuis plusieurs années et avec un soutien dépassant les clivages politiques, n'aient pas reçu meilleur accueil de la part de l'exécutif et des députés. C'est notamment le cas pour ce qui concerne le volet « assurance maladie », sur lequel nous partageons assez largement les orientations mises en oeuvre par Mme la ministre. Nous avons parfois le sentiment que certaines de nos propositions n'ont pas été réellement étudiées et qu'elles ont été écartées sans que soient véritablement recherchés les moyens d'apporter une réponse au problème posé. C'est pourquoi nous considérons, après la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, être parvenus au terme du dialogue utile sur ce projet de loi, comme l'a dit M. le rapporteur général. C'est donc en raison de désaccords fondamentaux sur la hausse de CSG et la politique familiale, mais aussi parce que les propositions que nous pourrions formuler à ce stade ne nous semblent pas pouvoir être prises en compte, que la commission des affaires sociales juge inutile de procéder à l'examen des dispositions restant en discussion et qu'elle demande au Sénat d'adopter la motion tendant à opposer la question préalable. La

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, à une époque où le citoyen se pose la question du rôle des élus, en particulier du Sénat, je regrette de devoir discuter de cette motion tendant

un accord. En première lecture, plus de 100 amendements ont été retirés. Souvent, après avoir écouté les arguments des uns et des autres, nous avons trouvé un consensus. Consensus en matière de prévention, tout d'abord, avec la hausse du prix du tabac, la taxe sur les boissons sucrées, l'extension de l'obligation vaccinale. Consensus en matière de simplification, ensuite, avec la fin du RSI son transfert vers le régime général, ainsi qu'avec la transformation du CICE en baisse pérenne de cotisations pour les employeurs. Consensus, en matière d'innovation, enfin, avec le développement de la télémédecine et l'amélioration du parcours de soins

Pour moi, choisir de ne pas examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale, même en nouvelle lecture, c'est nier notre rôle dans la procédure parlementaire. C'est nier notre travail d'analyse et d'approfondissement. C'est nier, enfin, l'importance des débats dans notre démocratie. On peut être en désaccord avec la politique du Gouvernement ; on peut critiquer la hausse de la CSG ou l'alignement des plafonds de la PAJE sur ceux du complément familial. Mais on ne peut pas dénigrer ainsi le débat parlementaire et s'en exonérer. Certes, l'Assemblée nationale a retoqué un certain nombre de dispositions introduites par le Sénat. Vous considérez, mes chers collègues, que le désaccord est si profond qu'il vaut mieux ne pas s'y pencher de nouveau. Il est vrai que, malheureusement, dès le premier soir de débat au Sénat, nous étions à 6 milliards d'euros supplémentaires en matière de dépenses. À la fin de l'examen, nous étions à près de 7 milliards déstructuration totale de l'équilibre budgétaire du texte ne pouvait être acceptée par le Gouvernement et la majorité présidentielle. Il n'est donc pas étonnant que l'Assemblée nationale ait pris en compte uniquement les propositions que je qualifierais de raisonnables qui ont émané de notre hémicycle. Je pense notamment à l'exonération de la hausse de la CSG pour les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, attestant d'une véritable et nécessaire prise de conscience de la spécificité du handicap. Je pense aussi à toutes les modifications apportées par le rapporteur général à l'article 11 et au RSI. Je pense enfin à l'exonération pour les véhicules de société roulant au superéthanol.

Pour ma part, je suis fier, avec le groupe La République En Marche, de soutenir ce projet de loi de financement de la sécurité sociale tel qu'il a été rédigé par le Gouvernement et amendé par l'Assemblée nationale, avec les apports du Sénat.

C'est aussi un projet de loi de financement de transition, en attente des grandes réformes sur la retraite, l'autonomie et le vieillissement en général, ainsi que sur la politique familiale. Je dois revenir encore une fois sur la remise en cause du mécanisme de la CSG pour les retraités et rappeler que l'effort que nous demandons est équilibré, à l'inverse d'un certain nombre d'autres décisions votées ici même, et qui continuent aujourd'hui encore d'affecter les plus fragiles de cette tranche de la population. Permettez-moi cette petite piqûre de rappel, mes chers collègues. En 2008, la majorité parlementaire avait voté la fin de la demi-part fiscale pour les veuves, avec une réduction progressive jusqu'à sa disparition totale en 2014. À cette suppression s'est ajoutée la fiscalisation de la majoration de 10 % des pensions des retraités ayant eu au moins trois enfants, jusqu'alors non taxée, décidée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.

C'est la seule possibilité pour notre pays d'avancer ; la seule possibilité pour notre système de protection sociale de subsister ; la seule possibilité de conserver un aspect protecteur et bénéfique pour les générations à venir.

l'opposition totale et résolue des membres du groupe socialiste et républicain aux deux points qui sont au centre de nos débats : la hausse de la CSG pour les personnes retraitées

Le scrutin est ouvert.